La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 5 octobre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire qui s'est réunie sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est parvenue à l'adoption d'un texte commun. La conférence des présidents, réunie jeudi 5 octobre, a décidé d'expérimenter des mesures de modernisation de la séance publique qui deviendront définitives en l'absence d'observations d'ici au début de l'année 2018. Par tradition, beaucoup d'annonces sont lues dans l'hémicycle, alors qu'aucun texte ne l'impose. La conférence des présidents a proposé d'en supprimer pour alléger la séance et de les remplacer par des courriels adressés à tous les sénateurs afin d'améliorer l'information de tous. Pour les nominations des sénateurs dans les organes du Sénat ou les organismes extraparlementaires, deux annonces successives sont effectuées en séance. La conférence des présidents a proposé d'en garder une seule indiquant le délai dans lequel la nomination sera ratifiée. Enfin, les conclusions de la conférence des présidents ne seront plus lues intégralement. Elles seront désormais disponibles pendant la séance et, en l'absence d'observation, elles seront considérées comme adoptées à l'issue de la séance. Nous expérimentons cette procédure dès aujourd'hui, avec les conclusions de la conférence des présidents réunie jeudi 5 octobre. Ces conclusions vous ont été adressées par courriel à l'issue de la réunion de la conférence et sont disponibles dans les couloirs d'accès à notre hémicycle et auprès des huissiers. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la suspension de la séance, avant les questions d'actualité au Gouvernement.- la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, cher Hervé Maurey, monsieur le rapporteur, cher Alain Fouché, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite, tout d'abord, adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes plus sincères félicitations pour votre élection ou votre réélection dans cette chambre haute du Parlement qu'est le Sénat. Je souhaite aussi vous exprimer tout l'honneur que j'éprouve en présentant aujourd'hui, au nom du Gouvernement, le premier texte de cette nouvelle session parlementaire soumis à votre approbation. Je sais que ce projet de loi, essentiel mais particulièrement technique, a été examiné dans des délais relativement contraints, qui sont notamment justifiés par l'urgence de ratifier ces deux ordonnances, j'y reviendrai dans un instant. Néanmoins, et malgré ce calendrier resserré, j'ai pu constater que les échanges en commission, jeudi dernier, monsieur le président, monsieur le rapporteur, ont été particulièrement riches. Je tiens à saluer le travail du rapporteur, Alain Fouché, qui a su s'emparer de sujets complexes que les élus locaux, dont je fais partie, connaissent bien. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a examiné, la semaine dernière, quinze amendements, dont onze ont été adoptés. visent à modifier des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale. Je pense néanmoins que nous pourrons facilement trouver un point d'équilibre. L'examen des amendements, tout à l'heure, me permettra de clarifier certains points. Pourquoi ce projet de loi est-il important ? Il permet de ratifier deux ordonnances fondamentales, prises le 3 août 2016, dans le cadre de la loi dite « Macron » l'une relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, pour reprendre la terminologie du droit communautaire, avec un objectif clair de simplification et de clarification des procédures ; l'autre permettant de réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public- c'est d'ailleurs sur celle-ci que les parlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, se sont plus particulièrement penchés une volonté d'associer davantage, en amont, les citoyens à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

le fruit d'une riche concertation au sein de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique menée par le sénateur et ancien ministre de la défense Alain Richard, dont je tiens à saluer le travail précis, de dialogue et

Cette concertation a permis d'obtenir un large consensus, que nous avons su conserver à l'Assemblée nationale et que nous allons conserver, j'en suis certain, au Sénat. Permettez-moi maintenant de revenir sur le contenu de ces ordonnances, en commençant, tout d'abord, par l'ordonnance n° 2016-1058 sur l'évaluation environnementale. Pourquoi cette ordonnance ? tout d'abord, de nous conformer au droit européen. La ratification de l'ordonnance permet, en effet, de conformer notre droit au droit européen, en transposant la nouvelle directive 2014/52/EU relative à l'évaluation environnementale des projets. Cette directive permet notamment de définir des critères d'évaluation pour mieux prendre en compte la santé, la biodiversité, le changement climatique, ou encore les incidences visuelles des projets sur le patrimoine Elle permet également de séparer les phases d'instruction et d'évaluation de certaines procédures environnementales à l'échelon local. Cette ordonnance à une simplification pour les porteurs de projets, tout en renforçant la protection de notre environnement. Je prendrai deux exemples concrets qui illustrent cet équilibre entre simplification et protection. D'abord, la simplification de l'étude d'impact que les élus locaux et les différents porteurs de projets connaissent particulièrement bien : les projets seront désormais appréhendés dans leur ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité des maîtres d'ouvrage. Cela signifie une étude d'impact en une seule fois sur chaque projet et non plus une étude d'impact par procédure.

Le développement de procédures dites au « cas par cas », ensuite, dans lesquelles on élève le degré d'exigence environnementale, mais en permettant à l'autorité environnementale de traiter ces demandes dans des délais plus courts, fait également partie de ces ordonnances. ordonnances. Monsieur le sénateur Ronan Dantec, en commission, vous avez parlé du rapport, que vous avez remis au nom de la commission d'enquête sur la compensation des atteintes à la biodiversité. Je tiens à vous préciser que le travail effectué à l'Assemblée nationale a permis de traduire,

J'en viens maintenant à l'ordonnance n°2016-1060 sur l'information et la participation du public. Pourquoi cette ordonnance ? Il s'agissait d'abord d'une réponse du gouvernement de l'époque- je la reprends à mon compte -à un changement de mentalité dans notre société qui s'est illustré avec la douloureuse crise, qui est d'ailleurs devenue un drame, de Sivens. Apprendre à perdre du temps en amont d'un projet ou d'une procédure pour ne pas en perdre ensuite » : cela paraît logique, mais nous n'avons pas toujours raisonné ainsi dans notre droit comme dans nos pratiques. Consulter en amont nos concitoyens permet, en effet, de lever les inquiétudes, de faire preuve de pédagogie, de dialogue, de répondre éventuellement à leurs doutes et à leurs craintes. Certes, Certes, la participation du public aux décisions environnementales n'est une nouveauté ni en droit ni en fait, et plusieurs textes nationaux comme internationaux l'ont déjà consacrée. Je pense notamment à la convention internationale d'Aarhus de 1998, de 1998, à la loi Barnier de 1995, qui a créé la Commission nationale du débat public, à l'article 7 de la Charte de l'environnement, adoptée en 2005, ou encore au Grenelle de l'environnement de 2010. Néanmoins, cette ordonnance permet de créer des droits nouveaux en réponse à une véritable demande de nos concitoyens, qui souhaitent davantage participer et même être associés à l'élaboration des décisions qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement. D'une part, les citoyens se sentent de plus en plus concernés par la protection de l'environnement. Ils développent clairement une conscience citoyenne, quelles que soient les idéologies et les philosophies autour de cette question. D'autre part, certains peuvent éprouver une forme de défiance

de veiller à ce que nos concitoyens puissent non seulement participer, mais surtout le faire au bon moment. Cette seconde ordonnance une réponse pour protéger l'environnement, mais aussi pour libérer et respecter les porteurs de projets, privés comme publics. publics. Elle permet en effet d'offrir aux porteurs de projets davantage de visibilité en amont de la procédure, et d'aller au-devant des problèmes pour les traiter le plus tôt possible.

premièrement, un droit d'accès aux informations pertinentes pour rendre la participation de chaque citoyen effective ; deuxièmement, un droit de demander l'engagement d'une procédure de participation dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons troisièmement, un droit à disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; quatrièmement, et cela est loin d'être neutre, à disposer d'un véritable suivi de la concertation et d'un retour- positif comme négatif -sur les observations qui ont pu être formulées par les participants au débat public. C'est une question de respect à l'égard du citoyen. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Ces droits nouveaux appellent naturellement de nouvelles modalités de consultation dans la forme et dans l'engagement. Première nouveauté : la CNDP, la Commission nationale du débat public, est obligatoirement saisie sur l'opportunité du débat pour les plans et programmes nationaux- on reprend la terminologie communautaire -soumis à une évolution environnementale là où, auparavant, seuls les très grands projets, c'est-à-dire d'un coût supérieur à 300 millions d'euros, étaient concernés.

sont actuellement rendus publics par les maîtres d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet qui indiquent leur décision de saisir ou non la CNDP. Ils informent ensuite la CNDP de la participation qu'ils prévoient. Grâce à l'ordonnance, les citoyens ont désormais un droit de saisine de la CNDP sur ces grands projets. Le seuil a été fixé à 10 000 citoyens de l'Union européenne ; c'est une innovation majeure, fruit du travail de concertation mené au Troisième nouveauté : ce droit d'initiative citoyenne est également ouvert pour les projets sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée percevant au moins

cher Alain Fouché, que vous êtes attaché au respect de la séparation de la loi et du règlement. C'est dans cet esprit que vous avez souhaité supprimer la mention d'un seuil de 5 millions d'euros pour la remplacer par un décret en Conseil d'État. Néanmoins, je tiens à rappeler le contexte qui a poussé les députés à inscrire dans la loi un seuil de 5 millions d'euros. C'est tout simplement le seuil permettant de prendre en compte des projets comme celui de Sivens, qui est justement à l'origine de ce texte destiné à apporter des réponses au drame que nous connaissons tous. Ce qui compte pour le Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n'est pas forcément que ce seuil soit inscrit dans la loi ou le règlement, mais qu'il s'établisse bel et bien à 5 millions J'espère donc que cette question de forme pourra être réglée entre les deux chambres du Parlement. Par ailleurs, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les différents échanges ont permis d'allonger à quatre mois, au lieu de deux mois, le délai offert pour exercer un droit d'initiative, ce qui constitue une avancée, notamment pour nos concitoyens les plus éloignés des décisions et des procédures publiques. Cet argument avait au demeurant été largement porté et défendu par les députés représentant des circonscriptions rurales. Vous avez fait le choix, monsieur le rapporteur, d'étendre ce délai de quatre mois aux collectivités et aux associations, dans un souci de cohérence. L'ancien maire et président de conseil départemental que je suis

les consultations pour les débats publics nationaux. L'ordonnance rend également possible le débat public national avec la saisine ouverte à 500 000 citoyens de l'Union européenne, à 60 députés ou 60 sénateurs, ou au Gouvernement sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples de ces politiques publiques. Ce seuil de saisine avait fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Je sais qu'un amendement du sénateur Guillaume Gontard

Le Gouvernement a cherché en permanence à être dans une démarche de simplification et d'alignement pour le citoyen, afin de ne pas avoir des seuils différenciés

Ces droits nouveaux ne bloquent pas, pour autant, les porteurs de projets, et c'est tout le fruit de l'équilibre de cette ordonnance. ordonnance. La CNDP veillera au respect des procédures et à la qualité de la concertation et des débats. C'est à la CNDP que le rôle d'organisateur des concertations a été donné. La CNDP occupe donc désormais donc désormais un rôle central dans ce dispositif. Ces nouvelles modalités de consultation nous ont obligés à davantage encadrer le rôle du garant qui sera directement désigné par la CNDP. Ces concertations ou débats devront répondre aux exigences d'un État moderne avec une nécessaire dématérialisation. Les collectivités territoriales et l'État

C'est une nécessité pour les porteurs de projets qui doivent aussi avoir de la visibilité ; c'est également une nécessité pour éviter tout contentieux. Aussi, la concertation préalable ne dépassera jamais trois mois et la durée de l'enquête publique est réduite de jours pour les projets ne relevant pas de l'obligation de l'étude d'impact. Concernant les délais, monsieur le rapporteur, vous avez fait le choix de revenir sur l'allongement de quatre à six mois du délai pour lequel l'illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut plus être invoquée par voie d'exception. Le délai de six mois avait comme mérite de s'inspirer de ce qui existe dans le code de l'urbanisme, permettant une harmonisation des procédures. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen des amendements. L'occasion m'est donnée devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, d'engager une réflexion collective, Parlement et Gouvernement, autour de la convergence du code de l'urbanisme, d'un côté, et du code de l'environnement, de l'autre. C'est quelque chose d'attendu, notamment par les élus locaux- je sais de quoi je parle. Là aussi, les éléments de simplification et d'alignement entre les deux codes sont les bienvenus. Avant de conclure, je tiens à préciser que je me suis engagé, à l'Assemblée nationale, le compte rendu fait foi, à mettre en place une première évaluation de ces deux ordonnances, afin d'en mesurer l'impact d'ici deux à trois ans et d'en tirer des modifications éventuelles. Nous créons des droits nouveaux. Il s'agit donc pour nous comme pour vous de voir de quelle manière nos concitoyens et les porteurs de projets vont s'en emparer. La parole est à M.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je suis très honoré d'inaugurer, comme vous, monsieur le vice-président, les travaux de notre assemblée pour cette nouvelle session. Je ne reviendrai pas sur le détail du contenu des deux ordonnances que le présent projet de loi a pour objet de ratifier : je vous invite à consulter le rapport, qui comporte toutes les précisions nécessaires. Ces deux ordonnances sont en effet techniques, mais elles touchent deux domaines très importants du droit de l'environnement, du point de vue tant de l'exigence qui doit être la nôtre en matière de protection de l'environnement, l'environnement, que de la nécessaire simplification des contraintes et des procédures pesant sur les entreprises et les collectivités territoriales. Je me bornerai donc à vous restituer les travaux de la commission et à formuler quelques observations. En ce qui concerne l'évaluation environnementale, que réforme la première ordonnance, la commission n'a pas apporté de modification substantielle. Il nous a semblé, en effet, que les travaux ayant précédé le travail de rédaction de cette ordonnance ont abouti à un équilibre acceptable. La simplification est réelle : elle se traduit concrètement par moins d'études d'impact pour les entreprises et les petites collectivités. Je souhaite cependant

Le premier concerne les inquiétudes de certains maîtres d'ouvrage, dans le secteur de la production d'énergie, quant à la nouvelle définition de la notion de « projet », qui risque de se traduire, selon eux, par une incertitude juridique, source éventuelle de contentieux. Le deuxième point concerne le coût des études d'impact et les délais qu'elles impliquent : sur ce sujet, l'ordonnance n'apporte pas de solution. J'ai été séduit, pour ma part, par l'idée avancée par notre collègue M. Alain Richard, ancien ministre de la défense, que j'ai pu consulter et dont je salue l'expertise, d'aller progressivement vers une « normalisation » de ces études. Enfin, monsieur le secrétaire d'État, disposez-vous d'une comparaison européenne un peu solide sur l'évaluation environnementale ? Plusieurs membres de la commission estiment indispensable d'être mieux informés et plus attentifs aux pratiques de nos voisins dans ce domaine. En ce qui concerne la seconde ordonnance, sur la participation du public, la commission a fait trois principales modifications. Elle a, tout d'abord, supprimé la fixation dans la loi d'un plafonnement du seuil de dépenses publiques à partir duquel un projet est soumis à déclaration d'intention et à droit d'initiative. Au-delà même du niveau de ce seuil, Au-delà même du niveau de ce seuil, le Sénat est attaché à ne pas empiéter sur le domaine réglementaire, car ce seuil doit être fixé par décret. Une telle précision dans la loi compromet également l'adaptabilité future du dispositif.

La commission a également harmonisé à quatre mois le délai durant lequel le droit d'initiative peut être exercé après la déclaration d'intention. Cette harmonisation me paraît tout à fait sage. Enfin, elle a ramené à quatre mois le délai durant lequel les vices de forme ou de procédure au titre d'une concertation peuvent être invoqués par voie d'exception lors d'un recours. Pour finir, mes chers collègues, je veux insister sur l'état d'esprit de notre commission. En vue de la séance, nous avons cherché avec les sénateurs concernés à intégrer de la meilleure dans le texte de ce projet de loi plusieurs modifications issues des propositions de deux rapports récents du Sénat, tous deux adoptés à l'unanimité : celui de M. Bonnecarrère, au nom de la mission d'information sur la démocratie, et celui de M. Dantec, au nom de la commission d'enquête sur la compensation des atteintes à la biodiversité.

les deux ordonnances qu'il nous est aujourd'hui proposé de ratifier s'inscrivent dans un long chantier de modernisation du droit de l'environnement qui s'est engagé sous la précédente mandature. Nous sommes évidemment tous favorables au fait de chercher à faire progresser l'évaluation environnementale et la participation du public dans les procédures, conditions incontournables à des débats apaisés. Nous sommes tous conscients, je crois, des difficultés dans la conduite des projets en France, à travers l'actualité régulière des mobilisations, voire des affrontements qui accompagnent certains grands projets d'aménagement, avec des risques réels de nouveaux drames humains, mais aussi à travers les dénonciations constantes, de colloque en colloque, des acteurs de l'éolien, par exemple, qui rappellent à juste titre que les durées d'instruction des dossiers sont doublées en France par rapport à l'Allemagne, soit huit ans contre quatre ans. Il y a donc aujourd'hui un intérêt commun entre les grands aménageurs et les associations défendant l'éolien citoyen à trouver des réponses aux blocages, par des processus d'évaluation globale des projets et de débats publics transparents où toutes les données sont sur la table. le secrétaire d'État, l'important travail de concertation réalisé en amont du texte discuté cet après-midi dans le cadre des groupes de travail sur la démocratie environnementale présidé par le sénateur Alain Richard, et sur la modernisation de l'évaluation environnementale présidé par Jacques Vernier. J'insisterai sur deux points précis de ces ordonnances qui me semblent particulièrement importants et novateurs. L'ordonnance sur l'évaluation environnementale complète le contenu de l'étude d'impact, et je souligne tout particulièrement l'introduction dans cette analyse de l'incidence du projet sur le climat le climat et sa vulnérabilité face au dérèglement climatique. Cela devrait aussi nous amener à évaluer certains projets d'infrastructures de transport au regard de leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'étude d'impact se fait également plus précise sur la biodiversité : il faut désormais décrire les mesures envisagées pour respecter la séquence éviter-réduire-compenser et définir plus précisément, point

qui va permettre de renforcer ce point. Par ailleurs, pour éviter que les concertations naturalistes ne surviennent après la première enquête publique, nous proposons que l'avis de l'Autorité environnementale soit complété par une réponse écrite du maître d'ouvrage à ses éventuelles objections dans le dossier d'enquête publique. C'est un point important,

du rapporteur : la rédaction actuelle nous semble fragile, car les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précisent que tout projet impactant sérieusement l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, même s'il est en dessous

ce droit reste très imparfaitement appliqué, et nombre de nos concitoyens se retrouvent souvent bloqués dans leurs demandes légitimes d'accès à l'information. C'est pourquoi je proposerai, d'une part, de créer un référé-communication pour faciliter un accès élargi aux informations environnementales et, d'autre part, de donner davantage de pouvoir à la Commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA, pour faire respecter l'application de ce droit à l'information. Il existe aujourd'hui des cas où, malgré les décisions de la CADA, l'État refuse encore de rendre publics les documents demandés, ce qui nourrit les colères et la détermination des opposants. Les ordonnances ne répondront pas à tout,

L'État et les maîtres d'ouvrage se sont souvent montrés frileux et méfiants sur ces débats, en pensant qu'ils nourrissaient la contestation. Notre analyse est inverse : c'est la faiblesse du débat qui nourrit avant tout les contestations.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté, et qui inaugure les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est donc un projet de loi de ratification de deux ordonnances prises à l'été 2016. Il s'agit de valider des réformes de diverses procédures d'information et de participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Le rapporteur a aussi proposé des amendements visant à ne garder dans la loi que les dispositions de nature législative, renvoyant pour le reste

Si le travail du rapporteur doit être salué, on peut regretter que les membres de la commission n'aient eu qu'un temps très bref pour s'approprier le texte et le rapport, et trop bref pour proposer d'aller plus loin. Vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur le secrétaire En effet, le sujet de la modernisation et de la simplification des procédures, notamment la consultation des citoyens, est inépuisable. Je relève dans ce texte au moins deux motifs de satisfaction. L'une des ordonnances prévoit que l'analyse des incidences sur l'environnement devrait intervenir le plus en amont possible, ce qui devrait mettre fin aux pertes de temps considérables que certains projets ont pu connaître par le passé, pertes de temps tellement pénalisantes pour l'économie d'un territoire ou même d'un pays. Il est aussi prévu une réduction du nombre des projets devant automatiquement- je souligne ce terme -être soumis à étude d'impact. On doit s'en féliciter. Il faut donc saluer l'objectif de simplification des procédures de consultation fixé dans ces ordonnances. Mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'un juste équilibre soit trouvé entre concertation avec le public et efficacité de la décision publique, entre protection de l'environnement et développement économique de nos territoires, entre principe de précaution et principe d'innovation. Ici, au Sénat, nous sommes tout particulièrement sensibles à la complexité et attachés à la simplification des normes et des procédures. En effet, les élus locaux que nous représentons, et que nous avons été- où sommes encore -pour la plupart d'entre nous, sont exaspérés par une complexité qu'ils ne comprennent souvent pas et qui est source de freins à l'initiative et aux projets, mais aussi de dépenses publiques, alors qu'on leur demande constamment de faire des économies. Par ailleurs, comme le rapporteur l'a souligné et comme je l'ai évoqué en commission, je pense que la rigueur des règles imposées devrait être mesurée par comparaison avec les procédures et règles applicables chez nos voisins européens. Il y va de la compétitivité de notre pays. Pourquoi serions-nous les plus tatillons ? Pour quel bénéfice ? Pourquoi la France est-elle le pays qui transpose le plus strictement les directives européennes, jusqu'à la surtransposition, reconnue, constatée et dénoncée par nos agriculteurs en particulier ? Que savons-nous des procédures et règles applicables chez nos voisins s'agissant de consultation des citoyens avant une décision environnementale ? Pas grand-chose ... Il me semblerait utile d'en faire une brève synthèse comparée ; ce serait même, à mon avis, un facteur de cohésion juridique des États membres de l'Union européenne. accélérée, utilisée sur ce texte déjà discuté à l'Assemblée nationale, ne permettra pas de le savoir. Il y aura, certainement, je l'espère, de nouvelles occasions de réflexion et de propositions plus approfondies

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte dont nous sommes saisis et qui porte sur la ratification de deux ordonnances marque

pour autant arrivés à une solution réellement satisfaisante ? Mon jugement sera mesuré. Je ne peux manquer de souligner que

au début ou en cours d'élaboration d'un projet, pour permettre une certaine conciliation des points de vue, ainsi qu'une prévention des conflits et des éventuels blocages,

je voudrais commencer par quelques mots de méthode. On ne peut pas se satisfaire des conditions d'examen de ce projet de loi. Les délais laissés aux parlementaires sont très resserrés. La commission s'est réunie pour sa constitution jeudi dernier et a examiné dans la foulée ce projet de loi. Quelques jours plus tard seulement, nous sommes réunis dans l'hémicycle pour son examen. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous réellement appréhender ces ordonnances importantes, puisque ce sont soixante articles du code de l'environnement qui sont impactés ? Cette procédure, cumulée à l'utilisation de la procédure accélérée, ne permet pas aux parlementaires d'effectuer correctement leur travail de législateur. Au final, nous ne pouvons corriger les dispositions de ces ordonnances qu'à la marge, sans revenir sur l'économie générale de ces textes. Pour cette raison, les sénateurs du groupe CRCE se prononcent régulièrement contre le recours aux ordonnances qui réduit le Parlement à une simple chambre d'enregistrement, puisque puisque ces ordonnances sont déjà en vigueur. Notre opposition est d'autant plus grande que cette habilitation a été votée lors de la loi Macron, loi à laquelle le groupe CRCE s'est opposé. Il existe, enfin, une contradiction évidente entre le fait de promouvoir la démocratie environnementale et la volonté de court-circuiter le Parlement. J'en viens au contenu. Sur la première ordonnance concernant la participation du public, si nous pouvons nous satisfaire de la volonté affichée d'améliorer le dialogue environnemental en amont de la prise de décision, les dispositifs préconisés paraissent particulièrement limités, voire lacunaires, et ce pour deux raisons principales. La première tient aux seuils de l'initiative citoyenne, manifestement trop élevés dans tous les cas de figure. Je ne prendrai qu'un exemple : recueillir l'approbation de 500 000 de nos concitoyens pour demander un débat public sur une réforme nationale semble bien inaccessible, encore plus dans des délais courts, fixés à quatre mois. Nous regrettons d'ailleurs, à ce titre, que notre amendement visant à diminuer de moitié ce seuil ait été déclaré irrecevable. La seconde raison tient dans l'absence d'obligation concrète du maître d'ouvrage de tenir compte des avis émis. On peut légitimement se demander s'il ne s'agit pas simplement de renforcer l'acceptabilité de projets contestés, voire contestables, et non de permettre, par l'implication citoyenne, d'améliorer et même de transformer le projet soumis à consultation. Vous avez d'ailleurs reconnu, monsieur le secrétaire d'État, que ces dispositions visaient simplement à « faciliter l'aboutissement de projets » ... Par ailleurs, les critères d'éligibilité des installations devant entrer dans le champ de saisine restent très restrictifs, notamment en ce qui concerne les seuils financiers. Pourtant, ni la convention d'Aarhus ni les directives européennes la déclinant n'autorisent à conditionner le niveau de participation citoyenne uniquement à des critères financiers. Il s'agit d'une vraie problématique sur laquelle les associations environnementales ont alerté les pouvoirs publics. Il existe des projets de faible ampleur financière aux conséquences très importantes sur l'environnement. La question reste donc posée d'une définition plus fine des critères pour permettre la participation des citoyens, laquelle est un droit constitutionnellement reconnu. Si l'Assemblée nationale avait amélioré le texte, le Sénat a fait le choix de revenir sur plusieurs avancées. Ainsi, des amendements avaient été adoptés afin d'abaisser la possibilité de saisine citoyenne pour les projets, programmes et plans à 5 millions d'euros comme seuil de dépenses publiques. Le délai concernant l'illégalité pour vice de forme ou de procédure avait été allongé à six mois. Le travail en commission au Sénat est revenu sur toutes ces améliorations. Nous le regrettons. Reste la question de fond. Dans un cadre exigeant et évident de préservation de l'environnement, quels seront l'impact et la portée réels de ce droit d'initiative pour nos concitoyens et pour la qualité de la décision publique ? Il faudra y revenir et évaluer ces dispositifs. Nous aurions pu aller plus loin, notamment concernant la question du référendum en matière environnementale- cette thématique est abordée dans le rapport présenté par Alain Richard. Les dispositions prévues paraissent donc timides et ne répondront pas à l'exigence souhaitée d'un meilleur partage des savoirs et des pouvoirs. La participation citoyenne semble si peu engageante pour les pouvoirs publics qu'elle risque même de s'avérer contre-performante en créant plus de frustration que d'enthousiasme. de la seconde ordonnance concernant l'évaluation environnementale, certaines de ses dispositions apparaissent clairement dangereuses. Il en va notamment de celles qui visent non pas à protéger l'environnement, mais à libérer les porteurs de projet, privés comme publics, de contraintes jugées excessives. Le Gouvernement se situe ici clairement dans la déréglementation, engagée et poursuivie par ses prédécesseurs au nom de la compétitivité coûte que coûte. Pour exemple, le passage d'une étude d'impact au cas par cas plutôt qu'automatique nous semble particulièrement problématique. La réduction des moyens dans l'administration risque, en effet, de laisser sans évaluation environnementale un grand nombre de projets, faute de temps et de moyens. Cela signifie que le respect du principe de non-régression du droit de l'environnement dépendra demain de la vigilance des services de l'État sur le terrain. C'est un risque que nous ne souhaitons pas prendre. Nous sommes donc, en l'état, défavorables à ces évolutions législatives. Pour autant, nous proposerons des amendements pour améliorer certains points de ces ordonnances. Nous espérons alors que le Gouvernement et la majorité sénatoriale sauront nous entendre.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la manière de décider a changé. Une décision est bonne non pas parce qu'elle l'est intrinsèquement, mais parce qu'elle est jugée bonne par ceux à qui elle a vocation à s'appliquer. L'aspiration des citoyens à s'exprimer directement et à être davantage associés à la prise des décisions publiques est incontestable. mes chers collègues, la légitimité et l'efficacité de la décision publique se voient de plus en plus contestées. Nous devons donc passer d'une légitimité de « position » à une légitimité de « décision », suivant la formule de M. Marcel Gauchet.

Comment, en effet, la démocratie participative peut-elle renforcer la démocratie représentative ? Comment mener à bien un projet d'infrastructure tout en veillant à la protection de l'environnement et à la consultation du public ?

connaîtrons plus tard de la ratification des deux autres ordonnances. Nous comprenons, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'enjeu politique qui existait en 2016 pour tenter de sortir de dossiers très douloureux que chacun de nous a en mémoire. Nous comprenons et partageons l'idée suivant laquelle, en consultant le plus en amont possible, il doit être possible de préparer et de dédramatiser la décision de réaliser telle ou telle infrastructure.

de valeur constitutionnelle, auquel M. le secrétaire d'État a fait référence dans son intervention préalable, mais aussi une directive européenne de 2003 qui avait déjà défini les modalités de participation, et que nous n'avions pas transposée. Rien, en résumé, ne fait difficulté dans le fond des deux ordonnances qui nous sont présentées, qu'il s'agisse de la définition plus précise des études d'impact-

Nous avons bien entendu, monsieur le secrétaire d'État, votre phrase, dont la presse s'était déjà fait l'écho, suivant laquelle il s'agirait de savoir prendre du temps pour mieux en gagner. Sur le principe,

La concertation est en effet respectable et nécessaire, mais la faisabilité de l'infrastructure l'est tout autant. L'objectif reste que notre pays soit capable de développer, d'aménager. Évitons l'exercice très français consistant à passer du tout l'un à tout l'autre ! Nous attirons votre attention sur l'équilibre prévu, qui consiste à mener plus de concertation en amont pour plus d'efficacité en aval.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Haute Assemblée examine aujourd'hui le projet de loi visant à ratifier deux ordonnances du 3 août 2016 relatives à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement. En effet, l'article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances dans le domaine du droit de l'environnement. À titre liminaire, je veux préciser que, selon nous, ces ordonnances sont essentielles. Je tiens, par ailleurs, à saluer l'implication du précédent gouvernement dans la rédaction de ces ordonnances,

Le travail que le Sénat fournit aujourd'hui respecte donc pleinement le principe de continuité républicaine, auquel nous sommes tous attachés dans cet hémicycle. hémicycle. Dès 2014, à la suite de la conférence environnementale, plusieurs groupes de travail se sont réunis. Cette riche concertation et les travaux menés en lien avec la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique présidée par notre collègue Alain Richard ont permis cette modernisation du droit de l'environnement. À l'issue de ce processus, un rapport a été rendu en mars 2015 par le président des groupes de travail, Jacques Vernier.

Selon nous, ces ordonnances vont d'autant plus dans le bon sens qu'elles reposent sur de grands principes, notamment l'article 7 de la Charte de l'environnement, laquelle a valeur constitutionnelle et consacre le principe du dialogue environnemental.

et l'ordonnance n° 2016-1060 tend à réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes D'une manière générale, nous ne pouvons que nous féliciter de mesures telles que le renforcement de la transparence, la participation plus facile du public à la concertation, notamment par la mise en place d'une plus grande dématérialisation, ou encore l'accroissement du rôle et des prérogatives de la Commission nationale du débat public.

de projets, plans et programmes, afin notamment de « mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ». Il s'agit donc bien de renforcer la concertation en amont, en amont « à un stade de leur élaboration, où ils peuvent facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public.

J'aurai l'occasion tout à l'heure de le présenter avec un peu plus de détails. Pour finir, je souhaite rappeler que ce projet de loi est d'autant plus important

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, quelques mots, au nom du groupe République et Territoires/Les Indépendants, sur ce premier texte de notre session ordinaire que nous examinons cet après-midi.

Il va de soi que, dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrai ni retracer l'état du droit avant les modifications proposées ni restituer en intégralité le travail accompli par notre excellent rapporteur Alain Fouché.

nationale. S'agissant de l'ordonnance relative à l'évaluation environnementale, je reprends la question que posent très bien les auteurs du rapport : de quoi parle-t-on ? De façon très simple, on peut dire que réformer le régime de l'évaluation environnementale, c'est s'inscrire dans une meilleure application du principe de prévention, la prévention consistant à empêcher la survenance des atteintes à l'environnement par des mesures appropriées, dites « préventives », avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité. On retrouve ce principe dans l'article 3 de la Charte constitutionnelle de 2004 qui impose à toute personne de prévenir les atteintes à l'environnement ou, à défaut, d'en limiter les conséquences. Notre rapporteur n'a pas proposé de modification substantielle de cette ordonnance. Il a très bien relayé des inquiétudes légitimes exprimées par certains maîtres d'ouvrage sur la nouvelle définition dite « englobante » de la notion de projet ; comme il le suggère, et nous y veillerons, il conviendra que les contours de cette définition puissent être rapidement précisés. Globalement, et nous y souscrivons, cette réforme permet une réelle simplification de l'évaluation environnementale, en particulier en allégeant des contraintes qui pèsent sur les petits projets et les petites collectivités. Dieu sait que notre assemblée est particulièrement attentive aux projets menés par les les collectivités de petite taille, qui regroupent l'essentiel du territoire de notre pays ! Le rapporteur a aussi proposé de réfléchir, sur la suggestion de notre collègue Alain Richard, à la normalisation des études pour en réduire les coûts. Nous sommes évidemment d'accord avec cette proposition et nous y souscrivons.

J'en viens à la seconde ordonnance, qui renvoie à la mise en oeuvre du principe de participation. Comme l'écrit le professeur Michel Prieur, la protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens.

débat public ou concertation préalable s'agissant d'un projet, enquête publique lors de la demande d'autorisation d'un projet ou d'approbation d'un plan ou programme. Cependant, chacun a en mémoire- Ronan Dantec l'a évoqué -les drames qu'ont pu provoquer différents projets la source de tensions et d'oppositions parfois violentes. Il faut donc renforcer et moderniser la démocratie environnementale, c'est bien l'objet de la seconde ordonnance. Là encore, le rapport est exhaustif et pédagogique, je vous y renvoie,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, premier texte de la session ordinaire, ce projet de loi de ratification d'ordonnances relatives au droit de l'environnement nous permet d'engager avec sérénité cette législature naissante. Depuis le premier Grenelle de l'environnement, le législateur ne compte plus ses efforts pour faire de la protection de l'environnement le préalable à toute politique publique responsable. Sur ce sujet, comme sur d'autres, le clivage droite-gauche me semble inopérant. J'ai d'ailleurs toujours dénoncé l'instrumentalisation de l'écologie pour des raisons partisanes. En cette année 2017, où tout le monde se doit d'être constructif ..., c'est dans un tel état d'esprit que je souhaite procéder à l'examen du présent projet de loi et de beaucoup d'autres- je l'espère ... Sans circonvolution, je veux donc dire que je voterai ce projet de loi de ratification. Comme mon collègue Gérard Cornu l'a précisé, vous ne trouverez personne au sein de notre groupe politique, Les Républicains, pour s'opposer à une réforme qui doit permettre de simplifier la vie quotidienne des collectivités territoriales et des professionnels, tout en assurant une meilleure association de nos concitoyens. C'est ce que réclament les citoyens et nos grands électeurs, comme je l'ai constaté dans mon département, la Mayenne, au cours de la campagne sénatoriale. sénatoriale. La première ordonnance relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes répond à la nécessité de simplifier le parcours des maîtres d'ouvrage, en prévoyant une étude d'impact par projet et non plus par procédure. Logiquement, cette réforme nécessite de renforcer l'étude d'impact qui devra désormais accompagner un projet tout au long de sa réalisation. Je souscris donc sans difficulté

peut apparaître, dans certains cas, superfétatoire. Toujours en ce qui concerne la première ordonnance, les projets seront répartis entre ceux qui sont soumis à évaluation environnementale de manière systématique et ceux qui le seront au cas par cas, et ce, afin de davantage recourir à ce second Toutes ces modifications sont appréciables pour les porteurs de projet qu'ils soient publics ou privés. Dernier point intéressant directement les collectivités, la nécessité de soumettre pour avis le document d'évaluation environnementale avant autorisation du projet à la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, en sus de l'autorité environnementale. Là encore, nous y souscrivons. S'agissant de la seconde ordonnance, portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, nous saluons, là aussi, l'esprit qui a présidé à sa rédaction. Cet esprit pourrait se résumer par la formule suivante : mieux associer nos concitoyens en amont pour gagner du temps en aval. Si nous analysons point par point les dispositions de cette ordonnance comme le fait le rapport d'Alain Fouché- renforcement de la concertation en amont des processus d'autorisation et modernisation de la concertation en aval, notamment par une dématérialisation accrue de l'enquête publique -, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Le seul accroc de cette parfaite harmonie réside, comme le rapporteur a eu l'occasion de le rappeler, dans la volonté de la majorité de marquer son territoire par rapport à une administration qu'elle doit déjà juger omnipotente. Si j'ai souvent eu l'occasion de constater que la volonté du législateur est reléguée au second plan lorsqu'il est question de publier des

son montant n'a jamais été évoqué par le législateur, parce qu'il s'agit manifestement d'une précision qui n'a rien à faire dans la loi, d'où le renvoi à un décret en Conseil d'État. Je suis donc favorable à la position du rapporteur de laisser le plafond à son niveau actuel- 10 millions d'euros -et non de l'abaisser à 5 millions. Je suis surtout favorable au respect de l'article 41 de la Constitution et je ne nie pas le fait qu'il est légitime de s'interroger sur le seuil optimal permettant la participation du public.

Surtout, ce texte doit nous faire comprendre que la complexité normative n'a rien à voir avec une haute exigence en termes de protection de l'environnement. Pour conclure, je plaiderai modestement pour une tâche qui, elle, ne l'est pas la rationalisation des articles liminaires du code de l'environnement, afin de redonner de la cohérence à une somme de dispositions qui cohabitent parfois difficilement les unes avec les autres. Je crois que, depuis l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, ce code a connu de trop nombreuses modifications et un travail analogue à celui que nous avons observé, en 2015, à propos du code de l'urbanisme serait le bienvenu. Les collectivités territoriales y seront attentives. Il y a donc beaucoup de travail en perspective en matière de simplification et je ne doute pas, pour l'instant, que le Gouvernement en soit conscient. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est avec un plaisir certain que j'interviens aujourd'hui dans l'hémicycle de la Haute Assemblée dans le cadre de la discussion du projet de loi ratifiant deux ordonnances du 3 août 2016 relatives à l'environnement. Ma qualité de nouvel élu de la République revêt pour moi un caractère solennel, particulièrement sur un sujet aussi sensible que celui de la participation du public. Le débat public constitue l'un des nouveaux liants de notre démocratie ; il implique la participation des citoyens bien au-delà des seules élections et doit être un facilitateur des décisions publiques. En outre, ces ordonnances viennent conclure plusieurs années de travaux : dès 2014, à la suite de la conférence environnementale, plusieurs groupes de travail se sont réunis pour moderniser le droit de l'environnement. Je suis attentif à quatre mesures phares. Premièrement, le renforcement du rôle et des prérogatives de la Commission nationale du débat public, organisme indépendant qui a su faire la preuve de sa pertinence et de son dynamisme et que je tiens à saluer. Pour ne rien vous cacher, j'en ai une une certaine connaissance, puisque j'y ai siégé quelques années comme représentant de l'Assemblée des départements de France. Deuxièmement, la création d'un droit d'initiative citoyenne pour l'organisation d'une concertation préalable à certains projets. Troisièmement, le renforcement de la transparence et une participation facilitée du public à la concertation, notamment par une plus grande dématérialisation. Quatrièmement, enfin, la clarification des procédures d'évaluation environnementale pour les projets, plans et programmes. exposé des motifs, qu'il s'agit de renforcer la concertation en amont « à un stade de leur élaboration, où ils peuvent facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public. » Cela vient faire écho au drame du barrage de Sivens, où le manque de dialogue et de concertation avait conduit à des blocages, des violences, puis à la mort d'un jeune manifestant. L'ordonnance n° 2016-1058 vise à modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et l'ordonnance n° 2016-1060 tend à réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Lors de son examen en commission, le projet de loi a fait l'objet d'une unanimité. Plusieurs amendements d'ordre rédactionnel ont été adoptés et d'autres sont venus préciser le texte, sans remettre en cause son économie générale. Il faut toutefois noter, avec un certain regret, que M. le rapporteur a supprimé le seuil de 5 millions d'euros à partir duquel est ouvert le désormais fameux droit d'initiative citoyenne. Il a en effet estimé qu'il fallait laisser au pouvoir réglementaire le soin de le fixer.

Ces amendements ont été rejetés, au motif qu'ils allaient au-delà du champ des ordonnances, mais certains d'entre eux ont toutefois reçu un large soutien sur le fond. J'aimerais aussi évoquer de manière positive deux amendements très récents.

afin de couvrir toutes les phases des projets d'infrastructure et pas seulement celles en amont. Il est positif de constater que, contrairement à sa première version, cet amendement fait la distinction entre le garant et le commissaire enquêteur. Dans une apparence de simplification, il était proposé de substituer le garant au commissaire enquêteur. Or le garant tire sa force de sa neutralité et du fait qu'il ne prend pas position, ce qui n'est pas le cas du commissaire enquêteur, qui doit rendre un avis. Enfin,

s'ajoute l'apparition de l'autorisation environnementale unique, je me tiens également à la disposition du Sénat pour mener ce travail sur les études d'impact, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un instant.

En effet, selon l'article 7 de la Charte de l'environnement, charte ayant acquis valeur constitutionnelle, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement L'ordonnance que nous devons ratifier aujourd'hui prévoit les conditions et les modalités de cette participation. Notamment, selon les termes du nouvel article L. 120-1 du code de l'environnement, la participation du public s'applique « dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence ». Nous estimons que limiter le principe constitutionnel de participation du public au respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique peut s'entendre, même s'il conviendrait d'apporter limiter le principe de participation au respect du secret industriel et commercial nous semble exagéré et ouvre la voie à de nombreux contentieux, car ce qui relève du secret industriel et commercial peut-être entendu de manière extrêmement large. Pour cette raison, nous proposons de supprimer cette mention, qui porte une atteinte trop importante en l'état à l'objectif affiché de renforcer la démocratie environnementale.

cette précision est un élément important du dispositif, qui assure un équilibre dans la mise en oeuvre de la participation du public. Elle vise à assurer aux maîtres d'ouvrage,

Il sera dans l'intérêt de tous que les informations pertinentes pour le public soient diffusées et que les éventuelles adaptations soient proportionnées aux enjeux économiques. J'ajoute que ce point n'a pas été soulevé lors des contacts que nous avons eus avec les différentes parties prenantes. Revenir sur cette disposition remettrait fortement en cause l'équilibre trouvé sur le texte pour les porteurs de projet. L'avis de

si vous menez un projet de zone d'aménagement concerté ou un projet de type ANRU dans un quartier

qui vont au-delà de ce qui était prévu par les ordonnances, pourtant à forte sensibilité environnementale, vous ne pourrez pas entamer la procédure de concertation prévue par le code de l'urbanisme, mais vous devrez vous adresser à la CNDP,

offre normalement le même niveau de garantie. Autrement dit, on ajoute des délais et on fait diverger les définitions des études de concertation. C'est la raison pour laquelle nous proposons de revenir au texte de l'ordonnance,

Monsieur le rapporteur, entre le code de l'environnement et le code de l'urbanisme en matière de concertation, pour un même projet. En substance, l'Assemblée nationale a choisi de faire prévaloir les dispositions du code de l'environnement, qui peuvent alors dispenser un projet des obligations de concertation au titre du code de l'urbanisme. La solution apportée par les députés nous semble pertinente, que les dispositions du code de l'environnement sont indiscutablement mieux définies que celles du code de l'urbanisme grâce aux ordonnances que nous examinons aujourd'hui. Par ailleurs, cette question ne se posera que dans des situations bien particulières : lorsqu'un même projet relève des deux régimes. Seule une partie de la quinzaine de projets qui sont soumis à la CNDP chaque année

amendement supprimerait cette faculté de concertation sous l'égide de la CNDP, alors que de tels projets gagnent à faire l'objet d'une discussion substantielle en amont.

Je soutiens bien sûr l'amendement n° 3 rectifié. En 2015, la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, présidée par notre collègue Alain Richard, avait mis en avant le sérieux et la qualité des concertations prévues par le code de l'urbanisme elles portent sur la révision de SCOT, la création des zones d'aménagement concerté, les projets et les opérations d'aménagement modifiant substantiellement le cadre de vie, les projets de renouvellement urbain. La disposition introduite à l'Assemblée nationale s'inscrit au contraire dans une logique de défiance, dès lors qu'elle ajoute une saisine de la Commission nationale du débat public. Cette saisine conduit à un temps d'attente qui peut déboucher ou non sur l'enclenchement d'une concertation relevant du code de l'environnement. Dès lors, cette dernière apparaît seulement redondante : il semble bien qu'il y ait une complexification. Nous entrons alors en contradiction avec un rapport sénatorial beaucoup plus récent, du mois de mai dernier, issu des travaux de la mission d'information à laquelle a fait référence notre collègue Bonnecarrère et que j'ai eu l'honneur de présider. La proposition n° 7 de ce rapport vise à simplifier les procédures applicables à la création d'infrastructures, en coordonnant davantage le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme. En commission, il a été dit contre cet amendement que seul un petit nombre de très grands projets serait concerné et qu'il était donc pertinent de mieux encadrer S'agissant des très grands projets, nous savons surtout qu'ils sont pleinement scrutés par tous les acteurs concernés et que la qualité du débat les concernant doit tenir au fait que ces acteurs se concentrent sur les nombreux enjeux de fond et non sur les chausse-trapes d'un grand nombre de procédures. Sur le fond, je crois utile de préciser ce que signifie pour moi la simplification, car j'entends les craintes qui s'expriment. Je vais prendre un exemple qui me tient à coeur, celui de l'artificialisation des terres agricoles. Je m'inscris pleinement contre cette artificialisation et je veux avoir les moyens de la combattre si un projet proposé n'est pas pertinent. Le terrain sur lequel je me place est bien celui de la pertinence du projet dans son environnement humain et naturel, telle qu'elle est discutée dans une concertation du type de celle prévue par le code de l'urbanisme. Si le projet ne me paraît pas pertinent, je veux le contrer pour une bonne raison, pour une raison de fond, et non pas parce que je pourrais avoir à ma disposition plusieurs procédures permettant de faire traîner les choses ou de soulever des vices de pure forme dont un magistrat devra préciser la portée. Pour moi, l'efficacité démocratique et la garantie des droits vont de pair avec la clarté des procédures que vise précisément cet amendement.

chacun un champ d'application clair et distinct- cette question est clarifiée par la jurisprudence depuis longtemps. Un projet soumis à une autorisation d'urbanisme, c'est une chose, un projet soumis à une autorisation d'environnement, c'en est une autre ! Aujourd'hui, cela a été vérifié en particulier par la Commission supérieure de codification, à laquelle nous sommes quelques-uns à participer, le degré de garantie d'information et de participation du public dans les deux procédures est équivalent.

Comme je m'y étais engagé lors de l'examen du texte en commission, je vous soumets cet amendement, qui répond à l'objectif visé par l'expérimentation proposée par notre collègue Philippe Bonnecarrère afin d'améliorer la continuité de la participation du public. En effet, j'avais rappelé que l'ordonnance comportait déjà un certain nombre de mesures contribuant à une meilleure continuité de l'information et de la participation pour un même projet, à la fois en amont et en aval des procédures. L'ordonnance prévoit notamment que la CNDP nomme un garant, chargé de la participation postérieure à un débat public ou à une concertation préalable décidée par elle jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Toutefois, cette disposition ne concerne que les projets relevant de la CNDP. Le présent amendement étend donc ce dispositif au projet hors du champ

lorsque les enjeux du projet le justifient. Il s'agit donc d'une solution concrète aux problèmes soulevés par notre collègue qui permet de compléter utilement l'ordonnance. Je tiens également à citer

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité

libéral, social et européen. Nous avons donc suivi avec beaucoup d'attention le récent discours du Président de la République, prononcé à la Sorbonne, sur l'avenir de l'Europe. Ses objectifs sont ambitieux : convergence sociale et fiscale, réforme des institutions, création d'une force commune d'intervention, etc. Nous approuvons ces objectifs,

Or il se trouve que les récentes élections au Bundestag vont sans doute contraindre la Chancelière allemande à former une coalition au sein de laquelle certains partis ont déjà annoncé leur scepticisme, voire leur hostilité, face à certaines de ces propositions.

ces obstacles pourront être levés ? Pouvez-vous plus précisément nous indiquer si vous avez déjà une idée de la feuille de route qui pourrait être suivie pour parvenir à ces objectifs annoncés ? La parole est à M. le Premier ministre. Monsieur

C'est un fait, ces élections ont consacré la victoire de la CDU, et, comme c'est souvent le cas en Allemagne, celle qui était désignée par le parti principal

la Sorbonne, a proposé à l'ensemble de nos partenaires européens de retrouver le sens de l'ambition collective qui avait été à l'origine de la construction européenne et d'avancer plus vite dans un certain nombre de domaines, à savoir le numérique, la zone Euro, la convergence sociale et fiscale ou encore la transition écologique. Deux jours plus tard, soit le 28 septembre, lors du sommet informel qui s'est tenu à Tallinn, tous les chefs d'État ou de gouvernement se sont accordés sur un constat au au fond évident : l'Europe doit se transformer si elle veut répondre à la promesse initiale ; elle doit se transformer, car tout le monde voit bien que son fonctionnement actuel n'est pas à la hauteur des enjeuxqu'elle doit affronter. Le chemin tracé par le Président de la République et l'ambition du projet qu'il a proposé ont été salués, singulièrement par la Chancelière Merkel et par l'Allemagne. Nous sommes donc tous d'accord sur l'objectif : il nous faut décider un nouvel horizon commun et remettre l'Europe en mouvement. C'est indispensable indispensable ! Je dirai que la discussion ne fait que commencer. Il était sain que la France fasse connaître sa position, utile qu'elle dise où elle voulait aller et quelles propositions elle formulait.

nationale, afin que l'on puisse avancer. La feuille de route qui a été fixée permettra, lors du Conseil européen des 19 et 20 octobre, puis lors du Conseil suivant des 14 et 15 décembre, de discuter entre les chefs d'État ou de gouvernement non seulement de ces propositions, mais aussi de celles qui ont été formulées par le président Juncker lors de son intervention voilà quelques semaines. Ce qui est lancé, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est une dynamique et c'est peut-être, à certains égards, une course contre la montre. Nous devons impérativement faire en sorte que l'Europe ne se satisfasse pas de la situation dans laquelle elle se trouve et qu'elle se remette en mouvement. C'est le sens des propositions fortes qui ont été formulées par le Président de la République et c'est, je l'espère, le début d'un débat auquel nous tous participerons,

Elles ont été sauvagement assassinées par un tueur radicalisé, aux cris et aux méthodes qui ne laissent aucun doute sur ses motivations. Nos pensées vont bien sûr tout d'abord à l'indicible tristesse de leur famille. Mais comment ne pas ressentir une colère profonde face à une telle abomination ? Même si nous avons tous conscience que le risque zéro n'existe pas en matière de terrorisme, interrogeons-nous sur le fait de savoir si le pire aurait pu être évité. Or force est de constater que la tragédie de Marseille n'aurait jamais dû se produire. Comment expliquer en effet qu'un clandestin, délinquant multirécidiviste, arrêté à sept reprises et sous sept noms différents, dont la dernière fois la veille du double meurtre, ait pu se promener librement sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille ? Comment ne pas être indigné lorsque l'on apprend que le tueur, au moment où il a tué, aurait dû être dans un centre de rétention ? Allez-vous enfin, monsieur le Premier ministre, sortir de cette hypocrisie consistant à demander au Parlement de voter toujours plus de lois, alors que leur application apparaît bien aléatoire ?

Pour moi, ce 1octobre a été un dimanche d'horreur. J'étais avec mes deux filles,

Je me suis immédiatement rendu à Marseille pour connaître les circonstances dans lesquelles s'était produit cet attentat.

Gilles, pour la réplique. Lutter efficacement contre le terrorisme passe, nous l'avons bien compris, par une dimension policière et judiciaire, mais la guerre que nous livrent les terroristes est aussi une guerre de sens, qui vise à conquérir les esprits. Le déni de réalité face au totalitarisme islamique est flagrant et paralyse malheureusement notre État. Il faut conclure ! Une violence extrême gangrène notre pays. Le combat est donc aussi culturel.

Le 23 février dernier, la Haute Assemblée adoptait une proposition de loi prévoyant le maintien des compétences « eau et assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes. Ce texte permettait de répondre aux attentes des élus locaux de nos territoires et, surtout, de laisser la liberté nécessaire dans l'organisation des compétences du bloc communal.

une fin de non-recevoir à cette question, alors que toutes les associations d'élus réclament un assouplissement de cette mesure prévue par la loi NOTRe. Quel mépris pour les élus ! Ce choix est particulièrement inopportun, puisqu'il dépossède les élus de nos territoires ruraux de tout choix, alors que, depuis des décennies, ils ont su mettre en place des solutions adaptées à la géographie et aux contraintes de leurs territoires. Ces choix ont permis d'assurer la gestion de ces compétences au prix le plus juste, dans l'intérêt de leurs habitants, dans l'intérêt de nos concitoyens. Pourquoi casser ce qui fonctionne ?

au sujet. Le Gouvernement a pensé, à la suite d'ailleurs de la demande de nombreux élus, qu'il fallait arrêter de changer les lois sans arrêt et que nous devions faire une pause dans la législation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur l'ensemble des compétences transférées par la loi NOTRe.

Le Gouvernement a voulu jouer cartes sur table lors de la Conférence nationale des territoires en mettant tous les sujets sur le métier, notamment la réforme de la taxe d'habitation, mais aussi l'investissement, qui participe à l'économie de nos territoires. Les collectivités locales ont besoin de visibilité sur leurs finances à long terme ; elles ont besoin de garanties sur la stabilité des dotations pour s'engager à investir. Les baisses unilatérales Les baisses unilatérales et uniformes de la dotation globale de fonctionnement dans la période précédente ont été mal vécues et ont laissé des traces. Par ailleurs, nous savons que cette logique partenariale commande d'assurer aussi de la justice pour différencier, dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les 319 collectivités les plus importantes et les autres, qui sont parfois aussi dans la difficulté. Il faut donc prévoir de la justice dans la redistribution, dans la péréquation. C'est l'un des objectifs du projet de loi de finances. au moment où le projet de budget met enfin un terme aux baisses de dotation aux collectivités locales, ce qui est inédit, pouvez-vous nous assurer que cette stabilité durera pendant tout le quinquennat ? Elle ne le

les crédits de la politique de la ville -augmenteront de manière très sensible pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Vous avez donc raison de dire que c'est la fin de la période du rabot unilatéral sur l'ensemble des collectivités.

financier avec l'État, les critères qui permettront de signer ce pacte. Pour répondre précisément à votre question, cet engagement vaut pour un an, bien évidemment, il faudra faire le point, toujours dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, sur les ajustements qu'il conviendra de réaliser à la fin de l'année fiscale pour voir si la maîtrise des dépenses, puisque c'est de cela et

qui sera le lieu de la concertation et du dialogue que l'État veut rétablir avec les collectivités territoriales.

est l'occasion d'exprimer de nouveau notre solidarité avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 6 septembre dernier, mon territoire, Saint-Martin,

l'ensemble des forces de secours qui se sont mobilisées pour intervenir et, dans le même temps, pour condamner les reproches qu'elles ont eu à souffrir quant à leur supposé manque de préparation et d'anticipation. Je le dis comme je le pense qu'ait été leur prépositionnement, il n'aurait rien changé à l'ampleur du phénomène et aux dégâts occasionnés. Lors de sa venue, le Président de la République a déclaré qu'il fallait faire vite, quitte à bousculer les règles. Ces paroles ne sont pas anodines, mais, comme dans toute situation difficile, le temps de réponse semble toujours trop long, alors que le travail reste colossal. Aussi, monsieur le Premier ministre, nous attendons non seulement des actions plus rapides sur la reconstruction et la réhabilitation des établissements et bâtiments publics, mais aussi des gestes forts en direction du monde économique et des populations les plus fragilisées. Enfin, il me plairait, si vous en étiez d'accord, d'être associé, comme les autres représentants du territoire, aux comités interministériels qui travailleront à la reconstruction. C'est ensemble que nous devons appréhender les nouveaux choix, en collaboration étroite et en confiance. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous aujourd'hui assurer aux habitants de Saint-Martin que la réponse de la France sera rapide et, surtout, proportionnelle à l'ampleur des dégâts subis ? La parole est à M. le Premier ministre.

psychologiques à certains égards, tellement l'ampleur de la destruction bouleverse la façon dont on voit l'endroit où l'on vit lorsque l'on a à subir un épisode climatique d'une telle intensité. La phase d'urgence, en partie seulement,

d'experts, qui sont venus le plus rapidement possible sur les deux îles afin d'apporter un soutien indispensable aux populations. Je vous remercie, monsieur le sénateur, de souligner le rôle exemplaire que ces renforts ont pu avoir.

Une fois la phase d'urgence passée, il faut reconquérir, d'une certaine façon, la vie quotidienne et revenir à une vie normale, pour autant que cela soit possible. Les commerces et les services ont recommencé à fonctionner les liaisons aériennes et maritimes commerciales ont repris, même si la reprise du trafic à l'aéroport Princess Juliana est plus lente que ce que l'on imaginait initialement. Les réseaux électriques et de télécommunications fonctionnent, eux, plus rapidement que ce que l'on redoutait initialement. Ils ont été réparés, pas complètement, mais à un rythme plus soutenu que ce que nous redoutions. Un certain nombre d'enfants ont pu faire une rentrée, dans des conditions qui sont évidemment très éloignées de la normale, mais ils ont pu recommencer les cours. À cet égard, j'ai eu l'occasion d'indiquer que je me rendrai à Saint-Martin pour la rentrée de la Toussaint, afin de vérifier les conditions dans lesquelles le plus grand nombre d'enfants pourront reprendre une scolarité normale dès cette date. J'irai sur place avec M. le ministre de l'éducation nationale. L'urgence,

On pense au tourisme, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'activités économiques dont le fonctionnement est complètement perturbé par la catastrophe. Aujourd'hui, ce sont plus de 4 000 salariés, sur l'île de Saint-Martin et sur l'île de Saint-Barthélemy, qui bénéficient d'un régime de chômage

Nous avons également mis en place un fonds d'urgence et mobilisons le réseau bancaire pour que les lignes de trésorerie des entreprises ne soient pas coupées et pour que ces dernières ne connaissent pas de difficultés bancaires. Nous avons en outre mis en place un moratoire en matière fiscale et sociale pour éviter que les entreprises et le système productif des deux îles ne se retrouvent dans une situation trop pénible. Nous devons maintenant penser et mettre en oeuvre la reconstruction. C'est la raison pour laquelle nous avons désigné un délégué interministériel, qui se tient en contact permanent avec l'exécutif de la collectivité territoriale. Je réunirai demain un comité interministériel de la reconstruction. Ce sera le troisième depuis le début du mois de septembre. L'objectif est de voir dans quelles conditions nous pouvons reconstruire les équipements publics et les réseaux

Tel sera le sens du travail du comité interministériel de la reconstruction et tel est le sens des échanges que j'ai eus avec le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Gibbes. Comptez sur le Gouvernement pour être extrêmement mobilisé sur ce sujet. l'État doivent être à la hauteur de l'enjeu que vivent aujourd'hui Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Je vous entends, monsieur le Premier ministre, mais il est toujours difficile de rassurer et de faire patienter celles et ceux qui ont été le plus impactés par le phénomène et qui s'inquiètent, à juste titre, de ce qui sera fait demain.

Dans le cadre du projet d'absorption d'Alstom par Siemens, le ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, a annoncé son intention de ne pas lever l'option d'achat des actions détenues par le groupe Bouygues dans le capital d'Alstom. L'argument invoqué par le ministre de l'économie est que « l'État a un rôle à jouer dans l'économie, mais ce rôle [ ...] n'est pas d'être assis sur un strapontin ... ». Cet argument désolant est irrecevable, car, en rachetant les actions détenues par Bouygues, l'État deviendrait le premier actionnaire d'Alstom avant son absorption par Siemens, ce qui lui permettrait de peser sur les choix stratégiques ultérieurs. M. Le Maire prétend que l'État serait plus efficace en se contentant de figurer dans un comité de suivi. Or, malgré la création d'un tel comité concernant le site de Belfort, les engagements pris sont loin d'être tenus. Par ailleurs, lors de l'absorption d'Alstom-énergie par General Electric, des promesses avaient été faites par le groupe américain à M. Macron, alors ministre, de créer un millier d'emplois en France. À ce jour, General Electric en a, en fait, supprimé autant, comme comme à Grenoble dernièrement, où notre collègue Guillaume Gontard a apporté son soutien aux salariés de General Electric Hydro. Une coopération étroite entre grands groupes industriels du ferroviaire est nécessaire, mais l'opération en cause n'est européenne que dans ses naïves intentions françaises, comme l'a écrit l'AGEFI. Il faut en finir avec ce dogme consistant à prétendre que, pour coopérer efficacement, il faut fusionner. Avec l'absorption d'Alstom par Siemens, près de 2 milliards d'euros, qui pourraient servir à autre chose, seront dilapidés en dividendes et primes de contrôle aux actionnaires, soit l'équivalent de huit années du budget de R&D d'Alstom. Tout se passe comme si le Gouvernement favorisait les intérêts financiers des actionnaires de contrôle du groupe Bouygues au détriment de l'intérêt national. Monsieur le Premier ministre, ne dilapidez pas les atouts stratégiques d'Alstom Nous vous demandons instamment d'exercer l'option d'achat de l'État sur les titres détenus dans Alstom par le groupe Bouygues et de suspendre l'opération annoncée pour ouvrir un large débat démocratique

un seul objectif : trouver une garantie pérenne pour l'emploi et pour notre économie. Ce sera désormais chose faite, monsieur le sénateur, avec le rapprochement d'Alstom

La nouvelle entreprise aura un actionnariat stable, avec un ancrage franco-allemand solide, un projet stratégique clair reposant sur des positions et des technologies reconnues.

La discussion sera animée, puisque des modifications du contenu de ces textes sont déjà annoncées, en matière de fiscalité immobilière, par exemple, alors même que le débat à l'Assemblée nationale n'a pas encore vraiment débuté. Parmi les priorités, nous examinerons la fiscalité, en particulier celle qui porte sur le patrimoine, car la justice contributive doit guider l'action de l'État. Nous analyserons si les moyens supplémentaires sont mis là où il le faut et si les économies proposées s'accompagnent des réformes qui permettront de ne pas sacrifier la qualité du service public. L'opinion publique y est sensible, les mobilisations de diverses natures le montrent ; c'est le Nous serons- lendemain d'élections sénatoriales oblige -particulièrement vigilants s'agissant des finances des collectivités territoriales. Nous veillerons aux modalités de la contractualisation et au fonctionnement du dispositif de bonus-malus, à la juste répartition des efforts entre collectivités et autres administrations publiques, sans parler de la réforme de la taxe d'habitation, qui ne doit ni réduire la capacité d'agir au plus près de nos concitoyens dans les territoires ni ajouter à la différence de moyens entre collectivités. Sur ce sujet, nous devrons disposer de toutes les simulations, que je ne manquerai pas de vous demander en ma qualité de président de la commission des finances. Sur les engagements européens, mon groupe a soutenu pendant cinq ans une politique qui conciliait redressement des finances publiques et préservation de la croissance. Peut-être cette approche fait-elle son chemin, puisque la dépense publique sera plus dynamique que vous ne l'aviez annoncé en juillet et même que ce que l'ancien gouvernement annonçait en avril. Vous proposez également, au nom de la croissance, un ajustement structurel inférieur à celui que demanderait une application stricte du droit européen. Sommes-nous soutenus par nos partenaires et par les autorités européennes dans cette lecture souple des règles ? Et, pour faire le lien avec notre débat de demain, la politique budgétaire du Gouvernement ... Il faut conclure ! ... place-t-elle notre pays en position de force pour faire évoluer la gouvernance de la zone euro ?

presque première des deux assemblées est de discuter, d'approuver, de corriger, voire, éventuellement, de rejeter, ce que je ne souhaite pas, le budget que nous proposerons. Les grands choix d'orientation de ce budget sont clairs. D'abord, nous tenons les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous les avons tenus, dès 2017,

et nous avons décidé, dès 2017, sans augmenter les impôts, de respecter les engagements européens que la France avait souscrits. Nous terminerons l'année 2017 avec un déficit inférieur à 3 %. Pour l'année 2018, nous présentons un budget conforme aux engagements pris par le Président de la République devant les Français, un budget qui innove sur un certain nombre de points. Je veux redire ici combien nous souhaitons mettre en place un mécanisme de maîtrise de l'augmentation des dépenses publiques des collectivités territoriales. Ce mécanisme passe non par une diminution de la DGF, mais bien par une discussion et un mécanisme

Il s'agit d'essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons, avec les principales d'entre elles, maîtriser cette progression de la dépense. Je le redis, nous souhaitons non diminuer les dépenses, mais maîtriser cette progression de la dépense. C'est un mécanisme nouveau. Comme tous les mécanismes nouveaux, il appelle des discussions. Il doit être

des interpellations dubitatives. Il serait probablement plus facile de faire comme nous le faisions avant, ou comme certains le faisaient avant, c'est-à-dire de diminuer au rabot la DGF. Tel n'est pas le chemin que nous prenons,

Si l'on ne discute pas de ce mécanisme dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, il n'y aura pas de discussions ! Et s'il n'y a pas de discussions, cela veut dire que cela se passera évidemment de façon brutale. J'invite l'ensemble de ceux qui

Comme chacun d'entre nous le sait, cela concerne les familles ayant au moins deux enfants à charge de moins de vingt ans. Déjà modulées en fonction des revenus lors du quinquennat précédent, les allocations permettent aux familles de bénéficier d'une aide financière mensuelle plus ou moins importante. Or les ménages les plus aisés pourraient bien se voir privés définitivement de ce droit- c'est en tout cas une proposition qui a récemment refait son entrée dans le débat public. Ce qui est gênant, c'est de revenir sur le principe même de l'universalité de ces allocations. Notre politique familiale est l'un des piliers de notre modèle social qui vient en soutien à toutes les familles ayant deux enfants. Évitons donc les caricatures grossières en opposant les foyers aisés aux plus modestes. La modulation a déjà marqué une évolution plus que symbolique en prenant en compte le niveau de ressources des familles, lors du quinquennat précédent. Je souhaite donc connaître, madame la ministre, les intentions du Gouvernement concernant ce sujet, qui touche un grand nombre de familles de notre pays.

Notre politique familiale est généreuse : 60 milliards d'euros en 2015. Cela représente 2,7 % du PIB. Elle se compose de modes de soutien diversifiés, dont la fiscalité, qui se cumulent entre eux au service des familles. Ce soutien public aux familles permet de maintenir leur niveau de vie et de concilier vie familiale et vie professionnelle. J'y suis très attachée, comme je suis attachée au principe d'universalité pour la sécurité sociale en général. La politique familiale a évolué ces dernières années, parce que la famille a évolué. On constate que certaines familles sont plus fragiles, notamment les familles monoparentales. C'est la raison pour laquelle le montant plafond du complément de libre choix du mode de garde sera majoré de 30 %. Cette mesure permettra à tous les parents qui élèvent seuls leurs enfants en bas âge d'être mieux aidés financièrement lorsqu'ils recourent à un assistant maternel, à une garde à domicile ou à une micro-crèche. Nous revaloriserons aussi deux prestations ciblées sur les parents isolés : l'allocation de soutien familial et le complément familial majoré.

le maintien des aides permettant de solvabiliser les modes de garde en préservant le libre choix des parents, de tous les parents, la création de places de crèche, en particulier dans les territoires sous-dotés. Nous assumons aussi un meilleur ciblage des aides monétaires destinées à soutenir les familles qui en ont le plus besoin, notamment les parents isolés et les parents à faibles revenus. Dans ce cadre, je souhaite entamer avec le Parlement et l'ensemble des acteurs un débat et une réflexion sur la politique familiale en général et sur les allocations familiales au service de cette politique. Il faudra prendre le temps, car la politique familiale ne se décide pas dans l'urgence. Vous l'avez dit, c'est un pilier de notre modèle social. Elle doit se discuter et être largement concertée avec tous les acteurs concernés. C'est la méthode de travail à laquelle je me suis engagée depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, et je m'y tiendrai. Madame la ministre, j'ai bien noté votre attachement à l'universalité des allocations familiales. Soyons effectivement fiers de notre politique familiale généreuse ! À quelques jours de la discussion du projet de loi n'ayez pas seulement une vision comptable de cet aspect de la politique familiale ! Si le taux de natalité dans notre pays est aujourd'hui supérieur à celui de nos voisins européens, c'est bien en raison d'une politique familiale historique. C'est en août 1946 qu'une loi a défini les quatre prestations de la branche famille de la sécurité sociale, dont les allocations familiales versées à l'époque sans condition de ressources à partir du deuxième enfant. Mon groupe, Les Républicains, est attaché à la politique familiale, à l'universalité de l'attribution des allocations familiales. La modulation qui s'applique depuis juillet 2015 suffit. Restons-en là ! Les enfants sont l'avenir de notre pays ! La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la européen. Madame la ministre du travail, je souhaite vous interpeller sur une décision préjudiciable que vous allez prendre pour les 126 maisons de l'emploi dans le cadre du projet de loi de finances pour Ce dispositif, mis en place par Jean-Louis Borloo dans la loi de cohésion sociale de 2005, a démontré depuis lors toute sa pertinence. Nombre de rapports d'évaluation en témoignent pertinence en matière de plan de formation, pertinence dans l'analyse des besoins des entreprises et pertinence, évidemment, dans la GPTEC, gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences. En clair, ces maisons sont des lieux reconnus d'ingénierie et de construction collective de l'emploi. Elles étaient initialement financées de manière paritaire par l'État et les collectivités. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les collectivités qui assument le budget des maisons de l'emploi à hauteur de 65 %. De 82 millions d'euros en 2007 à 21 millions d'euros en 2017, vous prévoyez un financement pour 2018 de 10,5 millions d'euros et de zéro euro pour 2019. Persévérer dans votre décision, c'est ne plus permettre à la ville de Bordeaux de porter les 215 000 heures d'insertion ouvertes auprès des jeunes de nos quartiers ! Persévérer dans votre décision, c'est empêcher, à Strasbourg, le PLIE, le plan local pour l'insertion et l'emploi, d'assurer la mobilité professionnelle vers l'Allemagne des jeunes en insertion. Et je pourrais vous citer bien d'autres exemples Force est de constater un nouveau désengagement de l'État sur une politique prioritaire. Est-ce ce signal, madame, que vous voulez envoyer, comme ministre du travail, à tous nos jeunes et à tous nos chômeurs de longue durée ?

Vous l'avez rappelé, les maisons de l'emploi ont été créées en 2005. L'idée initiale était de faire un guichet unique. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette date ; je pense notamment à la création de Pôle emploi en 2008. À ce moment-là, la notion de guichet unique s'est déplacée. déplacée. Les opérations de labellisation se sont arrêtées en 2009. Ensuite, tous les gouvernements, quelle que soit leur sensibilité, ont diminué peu à peu leur participation financière, considérant qu'il y avait des risques de doublons et qu'il fallait mobiliser toutes les forces ensemble. Je rappelle que la dotation était de 86 millions d'euros en 2009 et qu'elle a décru progressivement jusqu'à atteindre 21 millions d'euros en 2017. J'entends beaucoup de murmures sur les travées d'élus qui ont soutenu ces gouvernements. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Les maisons de l'emploi- il y en a 116 -ont, pour la plupart, évolué d'une façon complémentaire, laquelle consiste plutôt à aller vers les sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des bassins d'emplois. D'ailleurs, à ce titre, elles peuvent tout à fait bénéficier des financements

Compte tenu de la croissance qui repart, il y a des bassins d'emplois dans lesquels nous devons concentrer tous nos efforts pour permettre aux jeunes demandeurs d'emploi, aux jeunes décrocheurs, aux demandeurs d'emploi de longue durée de profiter de ces opportunités. C'est ce que nous ferons ensemble, et c'est mon souhait le plus cher

Il y a eu la vente de la branche énergie d'Alstom. Cela n'a pas été un succès- c'est un euphémisme ! Cela tourne au désastre Ma question est donc simple et directe : pourquoi refusez-vous d'acheter les actions Bouygues avant le 17 octobre pour que nous ayons un droit de regard sur ce projet de fusion ? Si nous n'avons pas ce droit de regard, inévitablement- Siemens a la majorité absolue et l'on connaît aussi la volonté de l'Allemagne de faire en sorte que son industrie soit la plus forte -, nous aurons de graves problèmes. Nous l'avons fait pour PSA. À l'époque, Pierre Moscovici avait proposé une entrée dans le capital de PSA. Les résultats sont là ! Arrêtons de brader les joyaux industriels et faisons en sorte de prendre ces actions pour avoir un droit de regard sur cette fusion

Nous croyons- c'est manifestement une différence entre vous et nous -à la construction européenne. Nous croyons à la réussite française dans le cadre de la construction européenne. Le nationalisme économique

coproduction industrielle pour faire un leader mondial de l'automobile ? Voilà ce dont on parle ! Si nous appliquions votre préconisation- ainsi que celle qui a été défendue tout à l'heure -, nous bloquerions immédiatement le rapprochement entre Siemens et Alstom. En effet, la condition de ce rapprochement pour faire un grand leader européen du ferroviaire, c'est justement que la France ne lève pas l'option. Alors, oui, nous pourrions avoir une approche spéculative

Monsieur le secrétaire d'État, votre angélisme me sidère ! Dans l'accord, Alstom conserve la possibilité de supprimer des emplois sur les sites en sous-charge, comme Belfort.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour le groupe Les Républicains. pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Dans le projet de loi de finances pour 2018, votre gouvernement s'apprête à concentrer le paiement de la taxe d'habitation sur seulement 20 % des Français à l'horizon de trois Ce que vous présentez comme une grande mesure de générosité, censée contrebalancer la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, pose de réelles questions de fond auxquelles vous n'avez pas donné de réponse. Tout d'abord, vous avez qualifié la taxe d'habitation de « mauvais impôt » et d'« impôt injuste ». Par quel miracle les défauts attribués à cet impôt ont-ils disparu pour justifier son maintien sur une partie de la population avant toute autre réforme ? Cette décision va encore accroître l'hyperconcentration fiscale qui pèse sur les classes moyennes, alors même que plus de quatre millions de ménages ont d'ores et déjà une taxe égale à zéro et que les foyers les moins aisés bénéficient d'allégements. Les contribuables qui gagnent plus de 20 000 euros par an et qui acquittent déjà par ailleurs l'impôt sur le revenu vont donc être les seuls à payer la taxe d'habitation. Ne pensez-vous pas que ce que vous présentez comme une mesure de justice apparaît en réalité très injuste ? Par ailleurs, une fois encore, ce sont les collectivités locales qui vont faire les frais de cette réforme. D'une part, elles nourrissent des inquiétudes quant au respect des services publics locaux- ce qui est gratuit n'a pas de valeur D'autre part, vous leur ôtez une part significative de leur autonomie fiscale en diminuant leur pouvoir de taux. Comment comptez-vous, dès lors, préserver cette autonomie, qui est garantie par la Constitution ?

Finalement, votre propos ne fait qu'illustrer les choix du Gouvernement : trouver des boucs émissaires, en l'occurrence, les collectivités locales, et concentrer l'impôt sur une infime partie de la population, celle qui vit du fruit de son travail, qui a pu acquérir un logement et qui paye donc par ailleurs la taxe foncière.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l'examen de l'article 2. L'amendement n° 18, présenté par M. Fouché, au nom de la commission,

en une année seraient susceptibles d'entrer dans le champ du droit d'initiative citoyenne si le seuil de 10 millions d'euros était maintenu. Cependant, le nouveau seuil de 5 millions d'euros a été supprimé en commission au Sénat au motif que cette précision venait empiéter sur le domaine réglementaire. l'ordonnance prévoyait initialement que ce seuil serait fixé par décret, sans en préciser le montant minimum. Si nous pouvons entendre cet argument d'un point de vue légistique et réglementaire, nous tenons à préciser qu'il arrive très souvent que la loi encadre le champ d'un décret. En outre, il nous paraît nécessaire d'ouvrir davantage ce droit d'initiative citoyenne afin de rendre le dispositif réellement pertinent et efficient tout en répondant à une attente sociétale forte.

sens, il est utile de préciser dans quel contexte s'inscrit cette discussion. L'ordonnance est incomplète et imparfaite sur ce sujet, puisqu'elle ne mentionne pas

La loi fixe les règles ou les principes, suivant les matières, mais, ensuite, c'est au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'application. Il est donc nécessaire de préciser la nature de l'opération qui est chiffrée.

Puisque, à 90 % au minimum, ce sont les collectivités territoriales qui seront assujetties à cette obligation, ce ne sera pas perdre du temps que d'assurer un minimum de concertation

à un décret en Conseil d'État l'ensemble des modalités de fixation du seuil.

au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur

ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordé sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant

je partage à la fois le propos de M. Richard et le propos de M. Cornu. Dans la logique de M. Richard, vous devez prendre un tout petit peu plus de temps pour traiter cette question par voie réglementaire en affinant la définition du seuil.

Nous proposons donc de limiter le rôle du préfet à l'examen de la recevabilité de la demande et du respect des critères fixés par la loi, sans l'étendre à des éléments d'opportunité. Tel est le sens de cet amendement qui aurait pour effet de rendre automatique la mise en oeuvre d'une concertation préalable dès lors que 20 % de la population du territoire concerné la demande. Voilà qui donnerait corps à ce nouveau droit qui va dans le sens de la démocratisation du dialogue environnemental.

de la convergence annoncée entre le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. Le premier point de l'amendement concerne la simplification.

Nous demandons, suivant le principe de convergence du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, l'application de la jurisprudence Danthony au code de l'environnement. Si une autorisation environnementale dite « unique

s'inspire des conclusions de la mission commune d'information sur la démocratie, dont vous avez été le rapporteur, mon cher collègue, et dont je tiens ici à saluer le travail. À titre personnel,

j'ai noté qu'il s'agissait d'une proposition de la mission commune d'information sur la démocratie, laquelle a rendu son rapport en mai dernier, et que certains de nos collègues y étaient très attachés. C'est la raison pour laquelle notre commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

des vices de forme ou de procédure au titre de la participation du public lors d'un recours contre une décision sur un projet. En commission, nous avons souhaité revenir à quatre mois, c'est-à-dire à l'équilibre défini par l'ordonnance. Invoquer pour seul motif une harmonisation par le haut avec le code de l'urbanisme nous semble insuffisant pour justifier la fixation de ce délai à six mois. Par définition, les dispositions de cette ordonnance vont créer de nouveaux risques juridiques pour les porteurs de projet.

? J'émets moi un avis très favorable, et je vais m'en expliquer devant vous. C'est davantage l'ancien président du conseil départemental de l'Eure qui

Il s'appuie sur une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle indique que la marge d'appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l'obligation qu'un projet fasse l'objet d'une étude d'impact dès lors qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d'effets avec d'autres projets, lequel ne peut s'analyser qu'une fois ces projets réalisés. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l'environnement, présidé par Jacques Vernier, à proposer l'introduction d'une clause-filet ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un petit projet, non visé par le régime de l'examen au cas par cas, mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L'objet de cet amendement est donc de mettre notre législation en conformité avec le droit de l'Union européenne, selon lequel les seuils ne sont qu'indicatifs, et d'ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif

à mettre en oeuvre cette clause en prévoyant que les projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement font l'objet soit d'une évaluation environnementale obligatoire

la France fait l'objet d'une procédure précontentieuse, puisqu'elle a reçu un avis motivé de la Commission européenne pour non-application de cette clause aux plans et programmes.

réponse figurera obligatoirement dans le dossier de l'enquête publique ou de la procédure de participation du public. En réalité, le maître d'ouvrage dispose déjà de la possibilité de modifier son étude d'impact afin de prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale avant le début de la procédure de participation du public.

le maître d'ouvrage doit réaliser une étude préalable comprenant une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets positifs et négatifs du projet sur cette économie et les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet, ainsi que les mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole. Cette étude complémentaire est adossée à l'étude d'impact.

Gontard. Par cet amendement, nous souhaitons pointer les contradictions entre le discours et le contenu réel de ces ordonnances. En effet, loin de la volonté exprimée en préambule d'améliorer la concertation et l'implication citoyennes dans la prise de décision pour les plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement,

Dans n'importe quel cas de figure, nous estimons qu'il n'est jamais bon signe de réduire le temps de l'information publique et de la concertation. Nous proposons donc de rétablir la durée de trente jours pour l'enquête publique.

de suivi des difficultés et des conflits, nous constatons que les enquêtes publiques peinent à remplir tout leur rôle, notamment sur deux points.

Comme l'on sait que l'enquêteur public va rendre un avis, le maître d'ouvrage essaie de le tirer par une manche pour qu'il soit favorable, et tous les opposants de le tirer par l'autre pour qu'il soit défavorable. En d'autres termes, l'enquête publique est instrumentalisée. L'intérêt du garant type CNDP,

assure la concertation, alors que l'enquêteur public, parce qu'on sait qu'il va donner un avis, est dans un camp et cristallise les difficultés. C'est pourquoi nous proposons d'expérimenter, dans le cadre du volontariat du maître d'ouvrage et de l'accord de la CNDP, l'hypothèse

les débats publics et les concertations relevant du champ de la CNDP portent aussi sur les modalités d'information et de participation ultérieures du public, et l'Assemblée nationale a étendu ces dispositions à toute concertation préalable. Après un débat public ou une concertation décidée par la CNDP, cette dernière désigne un garant chargé de veiller à l'information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Le garant ayant animé une concertation préalable peut être nommé commissaire enquêteur sur le même dossier. L'amendement n° 18, que nous avons adopté à l'article 2, permet d'étendre aux projets ne relevant pas de la CNDP la possibilité de nommer un garant chargé d'assurer la participation du public lors de la phase postérieure à la concertation préalable, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Comme je l'avais annoncé en commission, nous nous sommes efforcés de trouver, ensemble, une solution concrète à une question soulevée par la mission commune d'information sur la démocratie. Il ne me semble donc plus nécessaire d'instaurer une expérimentation spécifique, dont la mise en oeuvre exige la remise de deux rapports par le Gouvernement au Parlement, et qui revient, par ailleurs, sur le rôle même du commissaire-enquêteur. Considérant que

Les procédures de référé auprès du juge administratif sont des outils bien spécifiques, pour lesquels l'urgence, je le redis, est un élément central, qui justifie précisément la rapidité avec laquelle il est demandé au juge de statuer.

Les modifications proposées sont très larges, puisqu'elles ne sont pas spécifiques aux informations environnementales. Lorsque la CADA conclura au caractère communicable des documents réclamés, elle devra prescrire, dans son avis, le délai d'exécution de cette communication. Si ce délai n'est pas respecté, elle pourra sanctionner la personne responsable de cette communication.

Par ailleurs, la communication des documents administratifs ne relève pas du champ de compétences de notre commission. J'ajoute enfin que, sur le plan strictement rédactionnel, l'amendement fait référence à un article 18 indéterminé. Par conséquent, la commission a rendu un avis défavorable.

Avec cet amendement, nous voulons aller plus loin que ce que dispose le code de l'environnement dans sa version issue des ordonnances du 3 août 2016. En effet, si nous pouvons considérer comme une avancée significative le fait de soumettre à enquête publique les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, nous estimons que les exceptions prévues sont trop larges. Ainsi, il est indiqué que « cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier Nous comprenons pourquoi les installations soumises à l'octroi d'un titre minier ne sont pas concernées, puisque la concession minière est déjà soumise à enquête publique. Pour autant, à l'heure actuelle, les permis exclusifs de recherches minières ne sont pas, eux, soumis à enquête publique.

Pour cette raison, en espérant qu'aucune enquête publique ne soit à l'avenir nécessaire sur ce sujet, nous préférons, par prudence, inscrire dans le code de l'environnement une obligation de mener une enquête publique pour l'octroi

est déjà soumis à une procédure de participation du public. Il ne nous semble pas opportun de modifier ce régime au détour d'un amendement de séance, dans le cadre de l'examen selon la procédure accélérée d'un texte ne portant pas directement sur les sujets miniers.

La première créera ainsi un droit quasi fictif à la participation pour nos concitoyens, très éloigné des attentes exprimées. Nous sommes donc sceptiques sur la portée réelle de ces dispositions. Il faut savoir écouter, mais il faut aussi savoir entendre, et rien n'obligera demain les maîtres d'ouvrage à prendre en compte les observations et les critiques qui La seconde ordonnance passe d'une évaluation environnementale systématique à des évaluations au cas par cas. Certes, quand l'évaluation aura été décidée, elle sera efficiente. Mais que dire de tous les projets qui, du fait de ces dispositions, ne feront plus l'objet d'une évaluation, faute de temps et de moyens ? logement- les DREAL -que de dire qu'elles subissent de plein fouet les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements ! Nous avons voulu être constructifs et avons présenté des amendements. Aucun n'a été retenu. ne nous aura fallu que quelques heures pour modifier plus de soixante articles du code de l'environnement. Qui peut dès lors encore prétendre que la procédure des ordonnances respecte les prérogatives des parlementaires ? Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi de ratification. Personne